les réserves d'usage. Par lettre en date du 13 février 2019, M. Hervé Marseille, président du groupe Union Centriste, a demandé l'interversion de l'ordre d'examen des deux propositions de loi inscrites à l'ordre du jour de l'espace réservé à son groupe du jeudi 21 février 2019. Acte est donné de cette demande. L'ordre du jour appelle l'examen d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République islamique d'Afghanistan, d'autre part

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de la décision (UE, EURATOM) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les élections européennes sont un moment clé de la vie démocratique européenne. Pourtant, comme vous le savez et comme vous avez pu en faire l'expérience dans vos territoires,

Inverser cette tendance lors des élections européennes qui se tiendront entre le 23 mai et le 26 mai prochain dans les États membres, et le 26 mai en France, est un enjeu démocratique majeur. C'est aussi un enjeu politique essentiel au regard du fonctionnement même du Parlement européen. En effet, sur quelle majorité au Parlement européen le prochain président de la Commission européenne pourra-t-il par exemple s'appuyer ? C'est à chaque citoyen européen d'en décider et je sais que, légitimement, les opinions sont partagées dans cet hémicycle, mais je gage que nous nous réunirons au moins sur un point : personne ne peut se satisfaire de ce que nous avons trop souvent connu dans le passé, une campagne politique peu mobilisatrice et au fond bien plus nationale qu'européenne, une participation faible et une forme de cogestion entre les principaux groupes politiques du Parlement européen qui n'a peut-être pas été très stimulante pour les électeurs. Vous le savez, le Président de la République a souhaité redynamiser le projet européen. Cela passe par un renforcement de la légitimité, de la représentativité- sujet souvent débattu ces dernières semaines -et de la visibilité du Parlement européen. C'est dans cet esprit que la loi française du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen a été modifiée au mois de juin 2018, notamment afin de rétablir une circonscription électorale unique. C'est également dans cet esprit que les États membres ont entrepris, un an avant les élections européennes, de finaliser les négociations sur la modification de l'acte électoral de 1976, qui avait été lancée en 2015 par le Parlement européen. L'objectif de cette réforme était de rendre le processus électoral plus transparent pour les citoyens, mais aussi plus « européen », en renforçant les principes communs qui régissent les élections au Parlement européen. comment expliquer à nos concitoyens que les élections européennes obéissent à des règles aussi différentes d'un État membre à l'autre ? adopté le 11 novembre 2015, le Parlement européen a formulé des propositions ambitieuses pour renforcer les principes communs pour les élections européennes. Cela n'allait pas de soi, si l'on considère la grande diversité de traditions électorales au sein des États membres, tout comme la forte sensibilité de ces questions. De fait, les négociations au Conseil ont été difficiles et plusieurs propositions du Parlement européen particulièrement parlantes ont été rejetées, telles que l'instauration d'une date commune pour la tenue du scrutin ou la mise en place de mesures visant à permettre à l'ensemble des citoyens européens résidant à l'étranger de participer aux élections européennes. Les négociations au Conseil ont toutefois repris, après que les débats sur l'avenir de l'Union ont mis en lumière l'urgence de donner un nouvel élan démocratique à l'Union Elles ont permis d'aboutir à un accord entre le Conseil et le Parlement européen au mois de juin dernier. La décision modifiant l'acte électoral de 1976 a été adoptée par le Conseil des ministres le 13 juillet dernier, à Bruxelles. Il revient à présent aux États membres d'approuver cette décision selon leurs procédures constitutionnelles respectives. Cette réforme de l'acte électoral prévoit des modifications qui visent à renforcer les principes communs régissant l'élection au suffrage universel direct des membres du Parlement européen. Je précise, puisque c'est aussi une actualité européenne particulièrement brûlante, que même un Brexit sans accord serait sans incidence sur ces dispositions communes à tous les États membres.

S'agissant des députés européens eux-mêmes, l'article 1 de l'acte électoral est remplacé par un nouveau texte, qui précise que les membres du Parlement européen sont élus « représentants des citoyens de l'Union Cette modification, qui reprend les termes du traité de Lisbonne et s'inspire des parlements nationaux, vise à souligner la légitimité des membres du Parlement européen, qui représentent les citoyens de l'ensemble de l'Union européenne et non les citoyens du seul État membre dans lequel ils sont élus. Les États membres sont encouragés, dans un nouvel article 3 , à prendre des mesures pour que l'affiliation des candidats à un parti politique européen puisse apparaître sur les bulletins de vote, ce qui est d'ores et déjà possible en droit français, même si cette disposition n'a pas de caractère obligatoire. Là encore, il s'agit d'aider le citoyen à faire le lien entre son vote et l'action européenne de ses députés au Parlement européen. L'article 3 de l'acte électoral est également modifié, afin de rendre obligatoire la mise en place d'un seuil électoral dans les circonscriptions de plus de 35 sièges, compris entre 2 % et 5 % des suffrages exprimés- ce sujet a fait l'objet de discussions au sein de votre commission. Comme vous le savez, ce seuil permet de favoriser l'émergence de groupes politiques d'une taille significative et de faciliter ainsi le processus législatif au Parlement européen. Cette obligation doit intervenir pour les élections au Parlement européen de 2024, si la décision entre en vigueur avant les élections du mois Je rappelle cependant qu'en France la loi du 7 juillet 1977 fixe d'ores et déjà le seuil électoral à 5 % des suffrages exprimés. L'acte électoral révisé précise les dispositions à retenir pour la préparation et les modalités mêmes du vote. Il permet d'abord de mieux harmoniser le calendrier du dépôt des candidatures dans les États membres en prévoyant, dans un nouvel article 3 , une date limite pour le dépôt des candidatures, pour autant que la législation de l'État membre en prévoie une, au plus tard trois semaines avant le début de la période électorale. Cette disposition est donc cohérente avec ce que nous faisons en France, puisque la loi du 7 juillet 1977 fixe la date limite pour le dépôt des candidatures au quatrième vendredi précédant le jour du scrutin. Les États membres sont également encouragés à prévoir le vote par correspondance, le vote électronique ou le vote par internet aux élections européennes, ainsi et à mettre en place des mesures destinées à permettre à leurs citoyens résidant dans un pays tiers de participer à ces élections, comme le précise l'article 9 . En France, la loi du 7 juillet 1977 permet déjà aux citoyens français résidant à l'étranger de voter, lors des élections européennes, par procuration ou dans des bureaux de vote installés dans le réseau diplomatique et consulaire. Enfin, la décision qui vous est présentée prévoit, à l'article 9, que les sanctions contre le double vote seront renforcées, afin de s'assurer que les citoyens européens ne puissent pas voter dans plusieurs États membres à la fois. aux termes de l'article 9 , désigner une autorité chargée des échanges sur les données relatives aux électeurs et aux candidats, afin de faciliter l'échange d'informations entre les États membres. En France, le décret du 28 février 1979 charge l'Institut national de la statistique et des études économiques et le ministère de l'intérieur de transmettre aux autres États membres les informations relatives respectivement aux électeurs et aux candidats. La France prévoit par ailleurs, en cas de vote multiple, des peines qui peuvent aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et une amende de 15 000 euros. Je formulerai un regret, celui que le Parlement européen n'ait pas donné suite à la proposition qu'il avait initialement exprimée dans son avis du mois de novembre 2015, proposant la création d'une « circonscription électorale commune » dans laquelle les candidats auraient été élus sur la base de listes transnationales de chaque famille politique. La France avait défendu cette idée, qui aurait pu être mise en oeuvre pour un nombre limité de sièges et qui aurait contribué à une approche plus européenne de ces élections, ce qui est indispensable Le Conseil européen a dû faire le constat que cette idée ne pouvait être mise en oeuvre dès 2019. Il a néanmoins souhaité que les travaux se poursuivent dans la perspective des élections européennes de 2024. La France reste mobilisée et continuera à défendre cette idée. sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les grandes lignes de la révision de l'acte électoral. Elle représente au total une avancée européenne et une harmonisation progressive par le haut, qui entrera en vigueur lorsque l'ensemble des États membres l'auront autorisée. Je souligne que, compte tenu des normes dont nous disposons en droit français, l'approbation de la décision du Conseil n'appelle pas de modification des règles applicables aux prochaines élections européennes dans notre droit interne. La France, comme l'ensemble des États membres, est fermement attachée à ce que cette décision puisse entrer en vigueur avant les prochaines élections européennes. C'est pourquoi je vous demande d'autoriser l'approbation de la décision du Conseil du 13 juillet 2018. La parole

par un vote sur la décision du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct. Dans le monde difficile qui est le nôtre, l'Union européenne reste la seule voie possible si nous souhaitons conserver notre présence et notre capacité d'influence, à l'heure du retour des États-puissances et de l'affaiblissement de l'ordre international multilatéral. Pour avancer, le projet européen a plus que jamais besoin d'un nouvel élan, d'un nouveau souffle, et la légitimité démocratique de l'Union européenne en est le préalable.

dont on connaissait assez mal les limites et pour lesquelles il était assez difficile de nommer les députés élus. La décision du Conseil soumise à notre approbation poursuit cet effort d'harmonisation. Mme la ministre en a rappelé les principales dispositions : instauration d'un seuil d'éligibilité minimal commun à toutes les grandes circonscriptions, mise en place d'une date limite commune pour le dépôt des candidatures, plusieurs possibilités ouvertes aux États membres comme la faculté d'autoriser le vote en ligne, sous réserve d'assurer la confidentialité du scrutin. En tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, je regrette que le

modeste, puisque les dispositions obligatoires qu'il contient sont déjà intégrées dans notre droit interne et n'emporteront aucune conséquence juridique nouvelle. Cependant, tel n'est pas le cas pour l'ensemble de nos voisins européens ! Les modalités de scrutin étaient visiblement trop disparates entre les États membres pour permettre une véritable harmonisation dès les élections du mois de mai prochain.

Par ailleurs, une vingtaine d'États membres pratiquent le vote préférentiel, ce qui semble exclu en France et en Allemagne où le scrutin de liste bloquée est institué depuis très longtemps. La méthode retenue pour l'harmonisation des scrutins est donc celle, bien connue, Jean Monnet ! -, c'est-à-dire celle qui a prévalu pour la construction de l'Union européenne. Avec cette décision, les États membres franchissent un pas supplémentaire. Les négociations ne sont pas terminées pour autant ; elles seront relancées au cours de la prochaine législature

À titre personnel- car la commission ne s'est pas prononcée sur ce point -, j'espère qu'un consensus se dégagera sur des sujets importants, tels que la parité ou l'instauration des listes transnationales, qu'a mentionnée Mme la ministre. L'idée des listes transnationales figurait dans le rapport d'initiative législative adopté par le Parlement européen au mois de novembre 2015, avant d'être finalement retirée de la décision définitive du Conseil, faute d'accord. J'y suis pour ma part favorable : je pense que cela resserrerait le lien entre les citoyens et les institutions européennes et favoriserait le renforcement de la citoyenneté européenne.

pas moins qu'il faut faire progresser les idées. En conclusion, à l'heure où le populisme fait une percée aussi importante qu'inquiétante partout en Europe, tant au sein des parlements nationaux qu'au sein des exécutifs, il est de notre responsabilité d'apporter des solutions solides et fortes au lien qui s'est distendu entre les peuples européens et leurs représentants. La question des modalités électorales y participe. À cette fin, tous les pas vers une Europe plus souveraine, plus forte et plus juste sont les bienvenus. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter ce texte à la portée certes très limitée, mais qui est soutenu par la commission des affaires étrangères, de la défense

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, l'enjeu de ce projet de loi est très important, puisqu'il s'agit de la représentation de la France au sein du Parlement européen. Dans ces conditions, il est particulièrement regrettable que le Sénat ait initialement décidé de retenir la procédure d'examen simplifié

Cette façon d'agir, malgré les protestations que j'avais pu adresser à la commission des affaires étrangères, au président du Sénat et à différentes autres autorités de notre assemblée, caractérise un incontestable manque de transparence démocratique. Je remercie donc tout particulièrement Mme Assassi, présidente du groupe CRCE,

laquelle répartit les sièges de députés entre les États membres, que l'on prend soin de ne pas même évoquer dans les débats parlementaires, puisque le Parlement ne sera même pas consulté. Or le vice de constitutionnalité de l'une rejaillit sur l'autre. L'article 14 du traité de Lisbonne prévoit que chaque État doit avoir un nombre de députés européens « dégressivement proportionnel à sa population ». Comme l'indiquait la décision du Conseil du 28 juin 2013, qui a arrêté la répartition des sièges pour l'actuelle mandature, « chaque député du Parlement européen d'un État membre plus peuplé doit donc représenter davantage de citoyens

En 2018, lorsqu'il a fait ses propositions au Conseil des ministres pour la nouvelle répartition des sièges, qui sera mise en oeuvre au mois

Sur ce fondement, la décision prise le 28 juin 2018 par le Conseil a prévu que, si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, la France aurait cinq sièges supplémentaires. Le passage de 74 à 79 sièges respecterait alors l'obligation de proportionnalité dégressive. Toutefois, la même décision du 28 juin 2018 a prévu que, si le Royaume-Uni était toujours membre de l'Union européenne au moment des élections, l'ancienne répartition des sièges continuerait à s'appliquer jusqu'au départ effectif du Royaume-Uni. si le Royaume-Uni partait dans six mois, dans un an ou dans dix ans, on serait dans une situation évidente de violation du traité de Lisbonne. Madame le ministre, je vous ai interrogée sur cette problématique par une question écrite n° 7142 au mois de novembre 2018. Vous m'avez répondu, « si si le Royaume-Uni renonçait à sa demande de retrait, la décision du Conseil du 28 juin 2018 deviendrait caduque ». Madame le ministre, c'est de l'enfumage total et un mensonge à un double titre. et un mensonge à un double titre. Oh ! Oui, c'est faux ! Tout d'abord, rien n'indique dans la décision du Conseil du 28 juin 2018 que celle-ci deviendrait caduque en cas d'abandon du Brexit. Par ailleurs, les négociations avec le Royaume-Uni peuvent s'éterniser et durer pendant un an, deux ans ou plus : pendant toute cette période, nous continuerions à être dans une situation de violation du traité de Lisbonne. Pour toutes ces raisons et compte tenu des principes constitutionnels français, il me semble que les décisions du Conseil relatives aux élections européennes s'inscrivent dans une logique de violation du traité de Lisbonne et, indirectement, de notre Constitution. C'est pourquoi elles doivent être repoussées tant que la répartition des sièges entre les États membres n'a pas été définie dans un respect total, et non partiel, des termes du traité de Lisbonne.

de Lisbonne, qui pose un certain nombre de problèmes d'un point de vue démocratique : manifestement, la façon de concevoir la représentation dégressivement proportionnelle devient complètement abusive.

En application de cette disposition, pour la législature 2014-2019 du Parlement européen, c'est une décision du Conseil du 28 juin 2013 qui a fixé le nombre des députés attribués à chaque État membre. que cette répartition a été surtout dégressive et fort peu proportionnelle. En effet, on constate une véritable discrimination à l'égard des grands États,

qui, selon la Cour de Karlsruhe, n'a absolument aucune légitimité démocratique. Le tableau de la répartition des sièges pour la prochaine législature

Il est aussi savoureux de l'entendre s'intéresser au Conseil constitutionnel. Il est en revanche inacceptable d'entendre que le Gouvernement pratiquerait l'enfumage et le mensonge. Je tenais à réagir à ces propos qui, de mon point de vue, sont totalement inappropriés. Il est vrai qu'une partie

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre droit électoral, que nous avons récemment complété par la loi du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, rétabli une circonscription unique, converge vers la décision du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte électoral européen de 1976. Qu'il s'agisse du seuil minimal obligatoire pour l'attribution des sièges, du délai limite pour le dépôt des candidatures et de la « politisation » du bulletin de vote ou encore du régime de sanction du double vote, la France est dans les clous. Ce texte ne présentant pas de difficultés particulières, il aurait pu emprunter le cheminement discret de la procédure simplifiée. Aussi, sans entrer davantage dans le détail, le RDSE, qui s'enorgueillit de porter le projet européen dans son appellation même et qui a compté en son sein Maurice Faure, signataire du traité de Rome, approuvera le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui. L'objectif général d'une uniformisation des procédures électorales va dans le bon sens, celui d'une meilleure représentativité des députés européens. Néanmoins, dans le contexte d'une participation aux élections européennes en baisse depuis les tout premiers scrutins, nous pensons aussi que ce texte ne sera pas suffisant pour restaurer le lien entre les citoyens et leurs élus européens. C'est une difficulté que mon groupe avait déjà soulignée l'année dernière. En effet, nous avions alors soutenu le rétablissement de la circonscription unique, tout en rappelant la nécessité d'entreprendre un important travail de pédagogie sur le rôle croissant du Parlement européen au sein des institutions européennes. Nous avions déposé des amendements visant notamment à sensibiliser les jeunes Français au projet européen. Je rappelle en effet que les trois quarts d'entre eux ne se sont pas rendus aux urnes lors des derniers scrutins. Et je ne suis pas certain que la présence d'un drapeau européen dans chaque classe suffise véritablement à encourager l'esprit de citoyenneté européenne ! Quant à la proposition de listes transnationales dans le cadre d'une circonscription unique à l'échelle européenne, que le Président de la République soutient, mais qui est pour le moment repoussée, elle suscite chez moi les mêmes inquiétudes que chez certains de mes collègues. Il nous faut, en effet, trouver un système qui garantisse bien le pluralisme et la représentativité de tous les États membres. Je pense en particulier aux plus petits d'entre eux. Nous savons que le groupe de Visegrad, qui regroupe quatre pays d'Europe centrale- la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie -s'est farouchement prononcé contre l'année dernière dans une déclaration commune. C'est cependant un travail de réflexion que nous devrions poursuivre d'ici les élections de 2024. En attendant, au-delà du processus électoral, c'est sur l'idée même d'Europe que nous devons travailler. Le Président de la République l'avait rappelé en 2017, lors de son fameux discours de la Sorbonne, en invitant à « rendre l'Europe à elle-même et à la rendre aux citoyens européens ». Quand des crises et des défis se dressent face à l'Europe, il faut voir celle-ci comme un rempart, et non comme un bouc émissaire. Dans le monde ouvert d'aujourd'hui, on sait très bien que c'est l'union qui fait la force. N'oublions pas que seule une réponse collective a permis de gérer la crise de la dette et de traiter la crise migratoire. L'Europe est non pas la raison des problèmes, mais bien la solution aux grands défis. Le repli sur soi que certains prônent serait suicidaire. Il n'y a qu'à voir nos amis britanniques qui doutaient hier de l'Europe et qui doutent aujourd'hui de la sortie de l'Europe.

d'organiser un référendum national le 26 mai prochain, jour des élections européennes. Le RDSE est opposé aux mélanges des genres, ce qui ne fera que diluer les enjeux européens. Mes chers collègues, pour terminer, je reprendrai les mots de l'ancien président de la Grèce, Constantin Caramanlis, profondément européen : « Aveuglés par les différences de surface, ils n'ont pas su voir l'unité de la profondeur ». À l'approche de la campagne européenne, nous devons en effet en revenir aux fondamentaux de l'Union européenne, rappeler que la plupart des États membres partagent un socle de valeurs démocratiques et inciter les dirigeants à fixer rapidement un nouveau cap ambitieux et novateur à notre cher et vieux continent.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui approuve une décision du Conseil européen modifiant l'acte de 1976 portant élection des députés.

sont les objectifs louables de l'Union européenne : rendre le processus électoral plus transparent pour les citoyens, consolider les principes communs régissant les élections dans chacun des États afin d'en souligner le caractère européen

Nous ne pouvons qu'approuver ces mesures ou, plutôt, ces garanties. Vous nous demandez en effet, madame la ministre, d'approuver la convergence, l'harmonisation

moins souvent évoquée. La participation est le talon d'Achille de l'élection européenne : comment favoriser la participation de nos concitoyens le 26 mai et, plus largement, celle de l'ensemble de nos concitoyens européens ?

les ambitions que l'Europe peut porter, sur le réalisme de ses propositions et peut-être également, ce qui est plus délicat dans notre société, sur une vision de long terme tant l'Europe l'Europe se construit dans un temps long. Comment finalement surmonter, chers collègues, le paradoxe d'une Europe qui doute d'elle-même, alors qu'elle a franchi de nombreuses étapes ? Je rappelle qu'elle a créé un marché unique, une monnaie unique, unique, défini une charte des droits fondamentaux, développé l'espace Schengen, qu'elle s'est ouverte à des pays qui, pour les uns, ont pu y trouver la démocratie et, pour les autres, les conditions de l'indépendance et de la liberté, après l'effondrement du bloc soviétique.

Cette question nous confronte aussi, chers collègues, à la crise démocratique, à la crise de légitimité que traduisent nombre de prises de parole dans nos départements, dans le cadre du grand débat national. C'est une manière peut-être de vous dire, ou de nous dire, que tout est dans tout : à la fois la difficulté que nous avons à faire de la pédagogie sur les élections européennes, les débats, les contestations sur les éléments de la légitimité nationale et sur la manière dont, aujourd'hui, on

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « L'Europe, c'est l'espoir. Choisissez votre Europe » : tel était le slogan de la campagne pour les premières élections européennes au suffrage universel direct en 1979. C'était il y a quarante ans et, depuis, le Parlement européen n'a cessé de jouer un rôle de plus en plus important dans l'équilibre institutionnel de l'Union européenne, suggérant une progression irrésistible de la démocratie européenne. Pourtant, dans le même temps, la participation aux élections a connu une érosion progressive et systématique, pour atteindre des taux très faibles en 2009 et en 2014, respectivement 40,6 % et 42,4 %.

constante de légitimité et de reconnaissance. Alors qu'il est l'un des plus transparents dans ses décisions, le sentiment d'opacité est total, parce que les débats qui s'y déroulent échappent trop souvent aux populations. Il convient donc, à l'occasion de ces élections européennes, et sur la base des règles électorales en vigueur, de s'interroger sur ce désintérêt des citoyens. Trop souvent, nos concitoyens considèrent l'Europe comme illisible, obscure, éloignée, loin de leurs préoccupations du quotidien. Dans cent jours à peine, les Européens iront voter dans un contexte différent des scrutins précédents. Les questions d'immigration, du Brexit et de cybersécurité changent fortement le rapport des citoyens à l'Union européenne. Ces élections européennes doivent donc être, plus que jamais, une occasion de répondre à leurs attentes, qui sont fortes et nombreuses : les citoyens veulent une Europe qui les protège, une Europe sociale et solidaire, une Europe qui s'occupe des grands enjeux internationaux. Ces élections doivent être un moment fort de nos démocraties européennes, un moment clé pour l'avenir de l'Europe et pour ses citoyens, un moment qui doit mobiliser élus, citoyens, médias. Elles doivent être une occasion de répondre aux attentes des citoyens et de démontrer toute la légitimité du Parlement européen. Elles doivent être aussi l'occasion de dénoncer, comme vous le faites chaque jour, madame la ministre, les qui envahissent les réseaux sociaux pour décrédibiliser l'Union européenne.

après trois ans de négociations, les États membres et le Parlement européen sont parvenus à se mettre d'accord sur quelques critères énoncés dans la décision du 13 juillet 2018, sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui. Cette avancée est pour le moins modeste : les critères retenus changent assez peu la situation existante et sont, pour certains, non contraignants. Cela illustre aussi toute la difficulté de ces négociations, qui requièrent beaucoup de patience et de constance dans l'effort. Mais cette décision, même modeste, montre aussi, et avant tout, une volonté d'avancer et de faire du Parlement européen le coeur de la démocratie européenne. Elle va dans le même sens que le rétablissement de la circonscription unique. Il s'agit de renforcer la lisibilité de ces élections et de permettre un véritable débat national. Cette harmonisation de la procédure électorale dans les États membres, cette modernisation destinée à la fois à rendre cette procédure plus européenne, à renforcer la visibilité du Parlement européen et à renouer le lien entre l'électeur et le député européen, doit être saluée. Mes chers collègues, madame la ministre, il nous revient de faire des élections européennes ce grand moment de vie démocratique dont l'Union a besoin, et de faire du Parlement européen le coeur battant d'un projet européen porté par les peuples. Permettez-moi, pour conclure, de rendre hommage à celle qui fut la première présidente du Parlement européen, incarnation du courage et de la dignité, Européenne convaincue et dont l'image vient d'être honteusement vandalisée vrai ! Elle déclarait : « Se fixant de grandes ambitions, l'Europe pourra faire entendre sa voix et défendre des valeurs fortes : la paix, la défense des droits de l'homme, davantage de solidarité entre les riches et les pauvres. L'Europe, c'est le grand dessein du XXI siècle. » Soyons à la hauteur des paroles de Simone Veil et ne ratons pas le rendez-vous du 26 mai prochain ! La parole

l'acte électoral de 1976, lequel définit les grands principes d'organisation des élections européennes dans chaque État membre. Disons-le d'emblée, l'impact de ces modifications techniques sur notre droit électoral et sur l'organisation des prochaines élections européennes dans notre pays sera pour ainsi dire nul. Toutes les

Quant aux autres dispositions, elles demeurent optionnelles et, à l'exception notable du recours au vote électronique pour les Français de l'étranger, elles sont déjà appliquées. Dans ces conditions, le groupe Les Républicains ne voit pas de raison fondamentale de faire obstacle à ce projet Mais davantage que le contenu de ces propositions, ce sont les objectifs qui leur sont assignés qui retiennent l'attention. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, c'est animés de la volonté de « redynamiser le projet européen » et de lutter contre « l'érosion progressive et systématique » de la participation aux élections européennes que les États membres ont ont entrepris l'élaboration de ce texte suggéré par le Parlement européen. Au vu du contexte européen actuel, pour le moins tumultueux, de l'ampleur des défis auxquels l'Europe doit répondre, mais aussi de la désaffection croissante des citoyens pour le scrutin européen, ces objectifs apparaissent particulièrement pertinents.

sans doute de se contenter avec ce texte de viser une finalité plus modeste, à savoir le renforcement des « principes communs qui régissent les élections au Parlement européen, afin d'en souligner le caractère européen Il est en effet normal que les modalités d'organisation des élections européennes reflètent dans une certaine mesure le fait qu'il s'agit d'un scrutin à dimension continentale. À cet égard, je tiens à souligner le profond paradoxe qu'il y aurait à soutenir cette logique tout en accolant à ces élections la tenue d'un référendum. Dans une telle hypothèse, les enjeux européens ne pourraient que s'effacer derrière des enjeux nationaux de sortie de crise, ce qui serait une bien curieuse façon de souligner le caractère européen de la journée du 26 mai. Pour autant, je n'estime pas que le renforcement des principes communs qui régissent les élections européennes doive nécessairement aller jusqu'à l'instauration de l'éventuelle « procédure uniforme dans tous les États membres » qui est mentionnée dans le traité. Ériger cette notion en totem, comme le font certains, me semble à la fois vain et contre-productif. L'essentiel pour susciter l'adhésion des citoyens au projet européen ne réside absolument pas dans la standardisation de toutes les procédures électorales ou des jours de vote. Et si des règles communes à tous les États membres sont évidemment essentielles, elles ne doivent pas conduire à ignorer les traditions, les particularités et les sensibilités nationales, auxquelles les citoyens se révèlent parfois très attachés. Dans le domaine électoral comme dans les autres, l'Union européenne doit avant tout trouver la bonne distance et laisser aux démocraties nationales d'indispensables espaces de respiration. Évitons ce réflexe pavlovien qui consiste en matière européenne à confondre harmonisation et uniformisation. Et si cela est vrai en termes de procédures, cela l'est évidemment encore plus en termes politiques. Je fais ici référence à l'une des propositions phares du Président du Président de la République dans son discours de la Sorbonne, à savoir l'élection d'une partie des députés européens sur des listes transnationales. Malgré le revers considérable

Je souhaite réaffirmer notre opposition à de telles listes, car elles reposent sur une illusion, celle qu'il existerait un peuple européen. En outre, imaginer, comme Guy Verhofstadt l'a soutenu l'année dernière, que des listes transnationales pourraient et même devraient contribuer à le faire advenir relève tout simplement de la billevesée ou de la pensée totémique. Si les différents peuples qui composent l'Union européenne se sentent à l'évidence liés par une profonde communauté de destin- c'est d'ailleurs le sens même de la construction européenne-, ils ont avant tout pour cadre de référence la communauté nationale ou l'État-nation. Qu'on le veuille ou non, c'est au sein de cet espace public national que doivent s'organiser la vie et le débat politiques. Il demeure le creuset de la légitimité et de l'exercice de la démocratie, et ce ne sont pas les grandes envolées lyriques aux accents fédéralistes sur la « souveraineté européenne » qui changeront quoi que ce soit à cet état de fait. C'est une réalité tenace que l'on ne veut pas voir. À la différence d'une capacité d'action accrue des parlements nationaux dans le débat et le processus législatifs européens, par exemple l'instauration d'un droit d'initiative, voire d'un droit de veto, les listes transnationales ne seront en aucun cas capables de rapprocher l'Europe des citoyens et d'apporter une réponse au déficit démocratique de l'Union européenne. Il y a là une chimère aux couleurs européennes. Bien au contraire, de telles listes ne feraient que favoriser l'élection de députés européens « hors sol », et je dirais même « hors peuple », sans aucune prise avec les réalités du terrain ni aucun ancrage territorial, en d'autres termes, sans aucun lien avec les électeurs.

Il faut certes convenir que les huit circonscriptions interrégionales, trop étendues et ne correspondant à aucune réalité administrative, économique ou historique, étaient complètement vides de sens. Il faut aussi admettre que les députés européens élus dans ces conditions souffrent nécessairement d'un déficit démocratique et d'un déficit d'identification lié notamment à leur absence d'assise territoriale. Toutefois, la conclusion logique qui s'imposait face à ce constat aurait dû être l'introduction de davantage de proximité, par exemple en redécoupant les circonscriptions pour les faire coïncider avec des délimitations territoriales et électorales cohérentes. On a

en pire, que les circonscriptions interrégionales. J'entends déjà les déplorations vertueuses, le soir du scrutin, où l'on s'interrogera doctement sur le niveau de participation. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'argument selon lequel cette réforme permettrait de réduire l'abstention n'est que pure fantaisie. Il faut conclure, mon cher collègue. Par ailleurs, en prétendant donner plus de visibilité à la campagne européenne, on ne fera finalement que renforcer le poids des états-majors

Pour resserrer le lien aujourd'hui distendu entre l'Europe et les Européens, il s'agira avant tout d'élaborer, de confronter puis de mettre en oeuvre des projets politiques clairs et en prise avec les besoins et les aspirations profondes des électeurs. On peut toujours espérer Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, si notre groupe n'avait pas demandé ce débat, la convention qui nous occupe ce matin aurait été adoptée par la procédure simplifiée dans l'indifférence générale. Pourquoi un débat, me direz-vous, puisque la ratification de cette convention ne changera rien ? Elle réactualise celle de 1976, le Conseil européen l'a déjà adoptée et nous l'avons déjà transposée dans le droit français l'année dernière, en rétablissant notamment la circonscription unique nationale. Rien de neuf sous le soleil, donc, mais c'est bien tout le problème ! Dans trois mois, nous allons voter pour une élection européenne qui pourrait avoir de très graves conséquences sur l'avenir des peuples et des nations. Et que fait-on pour que les citoyens de notre pays soient saisis sérieusement des enjeux de cette élection ? Absolument rien ! J'entends dire qu'il faut faire ceci ou cela, mais nous sommes à trois mois de l'élection. Pourtant, ce n'est pas l'envie de débattre des Français qui fait défaut. J'entends parler d'indifférence, mais regardez ce qui se passe dans le grand débat national. Au demeurant, le débat de 2005 avait déjà montré l'intérêt des citoyens pour la question européenne. Pourtant, ce ne sont pas les signaux d'alerte qui manquent sur la très grave crise de confiance démocratique qui existe, non pas entre les citoyens et l'Europe, mais entre les citoyens de toute l'Europe et les politiques libérales obstinément poursuivies par les principaux gouvernements européens. Ces signaux ne cessent de se multiplier, à commencer par la chute régulière de la participation à l'élection européenne. L'Europe va au chaos, et tout continue comme avant. La question démocratique La question démocratique est au coeur de la crise politique que traverse notre pays, et au coeur de la crise politique que traverse toute l'Union européenne. Depuis des années, les grandes décisions sont prises en tenant à l'écart les peuples, contre l'intérêt du plus grand nombre, au seul service des grands intérêts financiers. Les résultats politiques de ce très grave déficit démocratique sont catastrophiques, mais où en parle-t-on sérieusement ? La France vient de rappeler son ambassadeur en Italie. C'est grave ! Le maire de Gdansk est assassiné dans un pays où le gouvernement attise la haine, s'attaque aux droits des femmes et à l'indépendance de la justice. C'est grave ! La démocratie est foulée aux pieds en Hongrie, où Viktor Orban vient de lancer sa campagne avec un discours qui réveille les échos des pires heures de l'Europe. C'est grave Les Britanniques ont quitté l'Europe et, à quelques semaines du Brexit, personne ne sait où l'on va. C'est grave ! L'émissaire européen de Donald Trump, Steve Bannon, a ouvert trois bureaux officiels à Bruxelles, Rome et Budapest pour coordonner la campagne des extrêmes droites européennes. C'est grave ! Mais où parle-t-on de cela sérieusement ? Les Français sont-ils saisis de ce débat ? Dans notre pays, les mobilisations sociales et le grand débat national mettent en exergue sur tout le territoire le besoin de services publics. Tout le monde le remarque. Mais, à Bruxelles, pas moins de quatre paquets de déréglementation sont de nouveau en débat, sans que ni les Français ni le Parlement national en soient saisis sérieusement- la question n'est d'ailleurs pas posée dans les débats publics qui ont lieu en ce moment. Et pendant ce temps, on privatise ADP, Engie, les barrages hydrauliques, et l'industrie européenne est soumise à de folles logiques concurrentielles. Oui, je le dis, il est fou de continuer comme cela, de ne pas débattre plus sérieusement de ces enjeux, de ne pas remettre au plus vite la souveraineté des décisions européennes entre les mains des citoyens, de ne pas saisir plus souvent et autrement le Parlement national de ces décisions qui engagent notre avenir. tout est fait une nouvelle fois pour brader le débat des élections européennes, pour l'expédier en quelques semaines sans permettre aux Français d'y intervenir réellement et consciemment, pour le caricaturer en le réduisant à un choix entre libéralisme et extrême droite, alors même que c'est ce choix tronqué qui conduit l'Europe au chaos. En France, la loi votée en juin dernier en application de cette convention comporte un seuil de 5 % qui déformera la représentation proportionnelle nationale, de même qu'une organisation scandaleuse des temps de parole pour la campagne des élections européennes. Le pluralisme est honteusement bafoué dans cette loi, et il conduira à des temps de parole sans aucun rapport avec la réalité des opinions parmi les citoyens de notre pays. Le déni démocratique continuera ainsi comme avant, comme si de rien n'était. Voilà pourquoi nous avons demandé ce débat, pour tirer une nouvelle fois la sonnette d'alarme, avant qu'il ne soit trop tard. Stoppez le déni démocratique, organisez autrement l'élection européenne, en permettant un débat réellement populaire, dans lequel l'option d'une Europe sociale, démocratique et écologiste retrouve le droit de cité et le temps de parole auquel elle a plus que jamais droit. Il faut conclure, mon cher collègue.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte n'est pas une révolution. D'ailleurs, le Gouvernement avait initialement proposé une approbation par voie simplifiée. Toutefois, grâce

de l'Europe, même si une implication plus importante des parlements nationaux serait utile pour faire converger un certain nombre de politiques qui, sans relever de la compétence communautaire, permettraient de faire mieux fonctionner l'Union européenne. l'Union européenne. Le fait que les critères démocratiques de Copenhague, au cours des dix dernières années, depuis la crise financière, se soient progressivement estompés au profit des critères de rigueur de Maastricht a profondément abîmé l'idée européenne, et c'est bien le risque majeur que nous affrontons aujourd'hui avant ces élections. Que dire de cette proposition, sur le fond ? Nous regrettons

qui proposait de créer une circonscription commune pour les citoyens de l'Union résidant dans un pays tiers, afin d'assurer à ceux-ci, de manière systématique et égale, le droit à une représentation au Parlement européen.

que, lorsqu'ils vivent hors de l'Union, ils puissent voter ensemble pour une représentation spécifique. Je voudrais aussi, madame la ministre, vous poser une question sur les manières de lutter contre les doubles votes.

nous permettra de transformer cette communauté de destin qu'est l'Union européenne en une réelle communauté de desseins, contrôlés et orientés par l'ensemble des citoyens,

n'a, dans mon souvenir, au cours des quarante dernières années, jamais demandé la fin de la proportionnelle pour les élections européennes. Je crois aussi devoir lui rappeler que cette même famille politique a été politiquement majoritaire au sein des institutions européennes

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative au délai d'intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, répondre à la situation migratoire à Mayotte est un impératif. C'est un impératif pour tous les Mahorais, qui connaissent mieux que tous les réalités d'une pression migratoire intense. C'est un impératif pour tous ceux qui tentent de rejoindre la France à Mayotte, que nous devons peut-être éloigner, mais envers qui nous avons un devoir de dignité. C'est un impératif, enfin, pour la République qui ne peut pas abandonner un de ses territoires, qui ne peut pas laisser courir le risque d'une sécurité menacée et de services publics embourbés. La réalité de la situation à Mayotte, c'est d'abord un chiffre : plus de 16 000 étrangers en situation irrégulière et que nous éloignons chaque année. Mayotte, c'est 260 000 personnes. Nous éloignons donc tous les ans l'équivalent de plus de 6 % de la population de Mayotte. À l'inverse, À l'inverse, on peut imaginer ce que représenteraient une machine grippée et des services qui ne pourraient plus suivre. Nous ne pourrions plus procéder à ces éloignements et la population mahoraise augmenterait chaque année en conséquence. Ce serait faire le lit de la misère, des tensions et de l'insécurité. Je le sais d'autant plus que nous avons été confrontés à cette situation pendant plusieurs mois en 2018, du fait de la suspension des réadmissions par les Comores de mars à novembre. Nous avons repris les éloignements depuis le mois de décembre à un rythme très soutenu, à raison de plus de 2 000 éloignements par mois. Cette situation, c'est celle que provoquerait l'application stricte de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Il y a donc urgence à légiférer. Il fallait agir vite, vous l'avez compris. Le Gouvernement et le Parlement ont donc travaillé pour agir en ce sens. commission des lois, cher Philippe Bas, vous avez permis que ce texte soit examiné dans les meilleures conditions et permis un dialogue constructif avec tous les groupes et le Gouvernement. Monsieur le rapporteur, cher Thani Mohamed Soilihi, vous vous êtes emparé de ce texte en amont, vous avez mené vos auditions en même temps que celles de la rapporteure à l'Assemblée nationale. Vous lui avez soumis un amendement qui est le fruit de votre travail et qui a été adopté par les députés. Vous permettez, en travaillant ainsi, qu'une réponse dans les temps, et adaptée pour Mayotte, soit ici proposée. Je voulais aussi vous en remercier. Je voulais enfin, plus largement, vous remercier pour le travail accompli afin de permettre l'examen de ce texte, pour répondre à l'urgence à laquelle font face les Mahorais. Durant la navette parlementaire du projet de la loi pour une immigration maîtrisée, le régime dérogatoire pour Mayotte en termes de saisine du juge des libertés et de la détention avait été supprimé. C'était pourtant bel et bien une erreur qui s'était glissée dans le texte, car ce choix ne correspondait à la volonté ni de l'Assemblée nationale ni du Sénat. Le texte que nous examinons propose le rétablissement à Mayotte du délai de cinq jours pour la première saisine du juge des libertés et de la détention. j'en suis convaincu, une mesure nécessaire pour maintenir un bon cadre juridique, solide et efficace, afin de permettre l'éloignement des étrangers en situation irrégulière qui tentent de s'établir à Mayotte. En métropole, le juge des libertés et de la détention est saisi par principe pour la première fois, dans un délai de quarante-huit heures après le placement en rétention. C'est un délai suffisamment bref pour garantir les droits de chacun, mais un délai suffisamment long, aussi, pour permettre de procéder à toutes les vérifications utiles et de prendre les mesures nécessaires.

et l'afflux de migrants, principalement venus des Comores, y est à la fois intense et constant. Mayotte, c'est donc une pression migratoire massive et permanente. Un chiffre pour l'illustrer : on estime que 48 % de la population présente à Mayotte est étrangère, et la moitié serait en situation irrégulière. Si nous appliquions le délai de quarante-huit heures, les conséquences seraient immédiates et probablement dévastatrices pour tous les services mahorais. Pour vous en convaincre, on peut imaginer simplement les conséquences d'un tel scénario. En réduisant de cinq jours à deux jours le délai de saisine, les juridictions devraient absorber dans un temps beaucoup plus contraint un nombre toujours aussi important de saisines. Pour suivre, il faudrait donc augmenter considérablement le nombre de personnels administratifs dans les juridictions et parmi les forces de l'ordre. L'impossibilité de traiter les demandes dans les délais conduirait immanquablement à mettre fin à la détention des intéressés. Le nombre d'escortes entre le centre de rétention administrative à Petite-Terre et le tribunal de grande instance, à Grande-Terre, c'est-à-dire sur une île différente, exploserait. Il faudrait donc une mobilisation permanente des forces de l'ordre pour escorter les retenus et une mobilisation permanente des personnels de préfecture chargés d'assurer le lien avec le greffe du juge des libertés et de la détention. Cela se ferait au détriment d'autres missions, au premier rang desquelles la lutte contre l'immigration clandestine. Ce n'est pas tout. Les conséquences sur le fonctionnement global de la justice à Mayotte, et donc sur la sécurité des Mahorais, seraient immédiates. Les personnels des juridictions et les juges des libertés et de la détention, les JLD, submergés par les demandes à traiter en quarante-huit heures, et déjà très fortement sollicités, ne pourraient plus se consacrer à d'autres missions. Je pourrais continuer, évoquer les conséquences sur les autres services publics, sur l'accès à la santé, aux ressources. Je pourrais aussi évoquer le signal très néfaste qui serait envoyé. choses en quelques mots, conserver cette mesure, c'est créer nous-mêmes l'embolie de la justice et de la sécurité à Mayotte. Alors, soyons pragmatiques et donnons à nos services publics les moyens d'accomplir leurs missions dans des conditions adaptées aux réalités locales. Le délai de cinq jours que nous examinons, lui, est parfaitement adapté à la réalité de la situation à Mayotte. Il est proportionné et ne réduit pas les libertés fondamentales des étrangers, qui peuvent toujours saisir le juge des libertés et de la détention et faire valoir leurs droits. Il ne réduit pas leurs droits en rétention et ne touche pas non plus la faculté du juge de procéder au contrôle de la mesure de placement. Mesdames, messieurs les sénateurs, la situation sécuritaire et migratoire à Mayotte est entre vos mains. Le 1 mars, en l'absence de vote dans les délais, le scénario catastrophe que j'ai dessiné pourrait devenir réalité. Nous pourrions rompre un équilibre en noyant sous les dossiers des services qui travaillent pourtant déjà d'arrache-pied et accomplissent, je le sais, un travail remarquable. Je sais que personne sur ces travées ne le souhaite et je peux vous garantir qu'il en est de même au Gouvernement. Cette proposition de loi permet de garantir à Mayotte un dispositif adapté ; saisissons donc cette occasion ! La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, nous sommes appelés à examiner la proposition de loi relative au délai d'intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte, adoptée par l'Assemblée nationale le 29 janvier 2019, après engagement de la procédure accélérée. L'objet de ce texte est technique et très circonscrit. Je n'y reviendrai pas longuement, car M. le secrétaire d'État nous l'a déjà exposé il porte sur le régime procédural de la rétention administrative à Mayotte, et il vise à corriger une erreur de coordination commise par l'Assemblée nationale lors de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Cette erreur doit être corrigée rapidement, avant le 1 mars, faute de quoi il y aura des conséquences néfastes pour l'efficacité des services en charge, à Mayotte, de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, auxquels je veux ici rendre hommage. À Mayotte, le JLD dispose en effet d'un délai maximal de cinq jours pour contrôler une mesure de placement en rétention, sur l'initiative du retenu, ou pour autoriser sa prolongation, à la demande du préfet, par dérogation au délai de quarante-huit heures applicable sur le reste du territoire. La proposition de loi qui vous est soumise vise donc simplement à conserver l'état du droit actuel à Mayotte, en y maintenant le délai dérogatoire un peu plus long dont dispose le JLD pour intervenir. Ce délai spécifique à Mayotte existe dans notre droit depuis 2017, et peut-être n'est-il pas inutile de rafraîchir les mémoires sur son origine. C'est sous le précédent gouvernement socialiste qu'il a été introduit, grâce à deux de nos collègues députés mahorais, à l'époque dans la majorité, soutenus par le rapporteur Victorin Lurel, et avec l'avis favorable de la ministre des outre-mer, De portée limitée, cette adaptation législative est parfaitement conforme à la Constitution, puisqu'elle permet de tenir compte des « caractéristiques et contraintes particulières » de Mayotte, comme le prévoit l'article 73 de notre texte fondamental. Vous connaissez en effet tous le contexte particulièrement difficile dans lequel s'inscrit la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. L'île subit depuis des années une pression migratoire exceptionnelle. La mission d'information menée en 2012 par MM. Jean-Pierre Sueur, Christian Cointat et Félix Desplan sur la mise en place de la départementalisation en faisait déjà le constat. Cette pression migratoire tient d'abord à l'attractivité économique propre du territoire- comme beaucoup de collectivités d'outre-mer, Mayotte a un niveau de vie moyen plus élevé que ses voisins mais il faut aussi prendre en compte le contexte géopolitique particulier et les liens historiques existant entre les îles de l'archipel des Comores. Les chiffres sont éloquents selon les premiers résultats du recensement de la population de 2017, près de 48 % de la population de Mayotte est de nationalité étrangère, ce qui constitue de loin la part la plus élevée de tous les départements français. On estime, en outre, qu'au moins la moitié des étrangers non natifs de Mayotte se trouvent en situation irrégulière. Ainsi, alors que l'île compte 256 000 habitants, le nombre d'étrangers en situation irrégulière oscillerait entre 60 000 et 75 000 individus. Les migrants, pour la quasi-totalité Comoriens venant des autres îles de l'archipel, effectuent leur voyage vers Mayotte grâce à des barques de fortune, les kwassa-kwassa, dans des conditions déplorables d'hygiène et de sécurité. Cet afflux constant de personnes en situation irrégulière contribue à désorganiser les services publics mahorais. Ai-je besoin de rappeler la situation de la maternité de Mamoudzou, qui doit accueillir près de 10 000 nouveau-nés chaque année ? Mayotte connaît ainsi une densité de population exceptionnelle, une urbanisation incontrôlée, la prolifération de l'habitat insalubre, et le développement de véritables filières d'immigration et de travail clandestins, aux dépens du développement socio-économique de l'île. Enfin, avec environ 20 000 reconduites à la frontière effectuées depuis Mayotte chaque année, ce qui représente près de la moitié des reconduites effectuées depuis l'ensemble du territoire national, et, en moyenne, 50 éloignements par jour, juridictions, associations, forces de police et services préfectoraux sont très fortement sollicités. Le maintien d'une disposition dérogatoire de portée limitée et purement procédurale à Mayotte répond ainsi à d'impérieuses nécessités opérationnelles. Dans un contexte de relations difficiles avec les autorités de l'Union des Comores, vers laquelle est reconduite la quasi-totalité des retenus en situation irrégulière, les éloignements doivent souvent être interrompus ou déplanifiés pendant quelques heures, voire plusieurs jours, incidents que le délai dérogatoire de cinq jours permet aujourd'hui d'absorber. La configuration géographique particulière de l'archipel de Mayotte doit également être prise en compte. Il n'est pas possible de multiplier les escortes entre le centre de rétention administrative de Pamandzi, situé à Petite-Terre, et le tribunal de grande instance, situé, lui, à Grande-Terre, sans détourner les forces de police de leurs missions. Enfin, ce texte ne modifie pas les garanties matérielles ou juridiques offertes aux étrangers retenus. Le centre de rétention administrative de Pamandzi, qui a ouvert en septembre 2015, leur offre des conditions sanitaires, de sécurité et d'accompagnement pleinement satisfaisantes, bien supérieures, même, à celles constatées habituellement sur l'île, comme le reconnaissent d'ailleurs, dans leurs récentes observations, les délégués du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. L'adoption de ce texte technique est donc nécessaire- j'espère que nous le voterons tout à l'heure, mes chers collègues mais, en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, ce sont surtout des moyens et des mesures concrètes que les Mahorais attendent aujourd'hui. Je me félicite de ce que l'État ait récemment consenti des efforts importants dans la lutte contre l'immigration irrégulière dans notre département des moyens techniques, tels que radars et vedettes, ont été débloqués pour l'interception des embarcations clandestines ; des renforts humains ont été déployés pour lutter contre les filières d'immigration clandestine et s'attaquer aux ressorts économiques et financiers du phénomène. Sur place, nous constatons que ces efforts commencent enfin à payer. Pour preuve, avec près de 2 400 éloignements réalisés au mois de décembre 2018, les forces de police ont retrouvé des niveaux d'efficacité inconnus depuis 2016. Il faut donc évidemment saluer ces avancées et le changement dans l'ampleur des moyens consacrés à ce problème. Cependant, je tiens aussi à insister sur le fait qu'il ne s'agit, pour l'essentiel, que d'un rattrapage, sur la base d'une situation extrêmement dégradée, qui a longtemps donné aux Mahorais le sentiment d'être abandonnés par l'État. Ces efforts méritent donc d'être non seulement poursuivis, mais amplifiés dans toutes leurs dimensions : les équipements et les renforts d'effectifs ne sont souvent pas assez nombreux, et ils restent encore sous-dimensionnés par rapport aux objectifs ambitieux affichés. Des moyens supplémentaires devraient être alloués à la lutte contre l'habitat et le travail illégaux, qui alimentent de véritables filières. Je n'oublie évidemment pas que la recherche d'une solution durable au problème passe aussi par la poursuite de la coopération diplomatique avec l'Union des Comores, pour favoriser le développement économique de toute la région et mieux dissuader ainsi les candidats au départ. Je souhaiterais aussi que les dispositions adaptant les conditions d'acquisition de la nationalité française à la situation migratoire particulière de Mayotte, introduites par le Sénat sur mon initiative dans la loi du 10 septembre 2018, soient accompagnées sur place de plus larges campagnes d'information. Je veux saluer, pour conclure, l'attitude constructive et pleinement respectueuse du rôle du Sénat qui a présidé aux échanges que j'ai eus avec le Gouvernement et avec mon homologue rapporteure de l'Assemblée nationale, Ramlati Ali. Nous avons ainsi, de notre commune initiative, modifié le texte initial par un amendement, adopté à l'Assemblée nationale, pour permettre au Parlement de disposer d'une information plus exhaustive sur les chiffres de l'immigration dans les outre-mer et à Mayotte, en particulier. Il s'agissait d'une demande récurrente, que je portais depuis de nombreuses années, et qui avait reçu l'appui du rapporteur, notre collègue François-Noël Buffet, lors de la discussion du projet de loi Immigration, asile, intégration.

Au bénéfice de ces observations, votre commission des lois recommande au Sénat une adoption conforme de ce texte utile et urgent. Une motion